Conformément aux articles 8 et 103 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe a été publiée. Cette liste sera ratifiée s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.

Annonce de la publication des listes des candidats à la commission des affaires européennes et de leur ratification sauf opposition dans le délai d'une heure.